La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du 18 janvier 2023 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation

L'importance du pastoralisme de montagne n'est plus à démontrer. Celui-ci contribue de manière essentielle, par son activité, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, ainsi qu'à l'emploi dans des zones très isolées. Dans le cadre de la future PAC, de nombreuses organisations, notamment des chambres d'agriculture, s'inquiètent des évolutions à venir. Les précisions qui ont été données L'exploitation collective des surfaces d'altitude, dites « d'estive », est en effet une particularité de l'agriculture de montagne. Elle fait intervenir, d'une part, les éleveurs transhumants et, d'autre part, les gestionnaires d'estive. Le premier pilier de la PAC de la PAC est destiné à soutenir les revenus des agriculteurs qui produisent de manière vertueuse. Les surfaces d'estive doivent donc être ventilées entre les différents transhumants pour l'activation et le paiement des surfaces Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir entendu la demande du monde pastoral concernant la répartition du versement de l'écorégime. Reste que le plafonnement des surfaces ligneuses un critère de chargement plancher qui serait fixé à 0,2 unité de gros par hectare est inadapté aux territoires pastoraux. Appliqué aux estives collectives, ce critère affecterait fortement le pastoralisme. Dans les seules Pyrénées, plus de 26 000 hectares seraient écrêtés, soit une perte d'aides de 7,3 millions d'euros par an. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, le Gouvernement entend-il limiter l'application de ce critère de seuil aux seules surfaces fourragères ligneuses des estives, ôtant du calcul toutes les surfaces fourragères herbeuses, afin de continuer à protéger l'espace pastoral ? La parole de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

hectare caractérise un type d'élevage extensif et permet aussi d'assurer un entretien minimal de ces surfaces. Ce critère de taux concernera uniquement les prairies composées majoritairement de ligneux, arbres, arbustes ou buissons

Or, quatre ans plus tard, l'article 14 de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 a assoupli cette contrainte, en autorisant les communautés de communes et les communautés d'agglomération à déléguer tout ou partie des compétences liées à l'eau, l'assainissement des eaux usées ou la gestion des eaux pluviales aux communes ou aux syndicats infracommunautaires existants au 1 janvier 2019. locale maintient l'échéance du 1 janvier 2026 pour le transfert, elle impose que les communautés de communes et les communes qui les composent organisent un débat sur la tarification des services publics de l'eau et de l'assainissement, ainsi que sur les investissements liés aux compétences transférées. Madame la ministre, les élus locaux ne veulent pas, à juste titre, que la compétence eau et assainissement soit gérée à l'échelle intercommunale. Les conseils municipaux souhaitent conserver ce levier, qui a aussi une dimension sociale.

Il faut tenir compte du fait que, dans les zones rurales, les coûts d'entretien par habitant des réseaux de distribution et de collecte ne sont pas les mêmes que dans les agglomérations. Comment une intercommunalité peut-elle gérer de façon efficiente ce type de difficultés ? Ne pas comprendre cette situation reviendrait à être hors-sol.

a, depuis lors, été transmis à trois reprises à l'Assemblée nationale : le 24 février 2017, le 6 juillet 2017 et, plus récemment, le 11 juillet 2022. Madame la ministre, je souhaiterais connaître la position du Gouvernement sur cette proposition de loi et savoir si vous soutiendrez ce texte lors de son examen à l'Assemblée nationale,

000 l'assainissement collectif. Cet émiettement est un facteur d'inefficacité et de dilution de l'ingénierie, qui fait obstacle à la bonne connaissance du réseau, à son rendement et à sa bonne gestion. Le passage à l'échelon intercommunal permettra de disposer de services ayant la taille critique pour assurer une bonne maîtrise et la performance des services d'eau et d'assainissement. Il permettra d'assurer un service durable, à un coût maîtrisé pour les usagers, par la création d'économies d'échelle mutualisation efficace des moyens techniques et financiers. Cette mesure de transfert n'est d'ailleurs pas nouvelle. Elle a déjà fait l'objet de nombreux ajustements, afin, d'une part, d'adapter les textes aux réalités concrètes

Deuxièmement, la loi Engagement et proximité a ouvert aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération la possibilité de déléguer, par convention, tout ou partie de ces compétences à l'une de leurs communes membres. la loi 3DS autorise les EPCI à mobiliser plus facilement leur budget principal, pour financer les compétences eau et assainissement, et prévoit l'organisation, dans l'année qui précède le transfert obligatoire, d'un débat préparatoire avec les communes membres. C'est pourquoi le Gouvernement ne souhaite pas revenir en arrière sur les transferts des compétences eau et assainissement. À l'occasion des travaux de planification écologique,

sur lesquelles elle souhaite se porter candidate, notamment au regard de la complexité technique de gestion de ces ouvrages. Selon les règles bien établies pour les transferts, le droit à compensation des collectivités territoriales bénéficiaires du transfert sera calculé à partir d'une moyenne des dépenses constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert, pour les dépenses d'investissement, et sur une période de trois ans, pour les dépenses de fonctionnement. Le décret qui doit fixer ces périodes de référence en application de l'article 150 de la loi 3DS est en cours de signature. Le 16 novembre 2022, il a été soumis pour avis à la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), composée à parité d'élus et de représentants de l'État, et a fait l'objet d'un avis favorable à l'unanimité. Concernant la méthode de calcul du droit à compensation, un certain nombre d'informations ont déjà été communiquées, les préfets, aux collectivités territoriales dès le mois de juillet 2022, par une instruction du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

des collectivités territoriales intéressées par le transfert de compétence. Enfin, la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) prépare actuellement, en lien avec la direction générale des collectivités locales, locales, un projet de décret fixant les modalités précises du calcul du droit à compensation, sans s'écarter des principes fixés dans la loi. Les assiettes de dépenses relatives aux différents postes de prestations seront ventilées selon les unités d'oeuvre correspondantes. Ainsi, les dépenses de chaussées seront ventilées au prorata des surfaces de chaussées, les dépenses d'ouvrages d'art au prorata des surfaces d'ouvrages d'art, etc. Une décomposition du réseau routier en trois grandes catégories- routes bidirectionnelles, routes à chaussées séparées, routes à chaussées séparées à fort trafic -et la prise en compte des particularités des routes à hiver rigoureux, ainsi que des itinéraires de montagne, permettront de déterminer un droit à compensation au plus près des besoins réels de l'infrastructure,

Moscovici, a déclaré : « Il ressort d'une façon générale et unanime que le sort de l'avenir des communes semble décidé. La dotation globale de fonctionnement, la célèbre DGF, va devoir aller vers les intercommunalités en sa totalité. On se dirige donc vers une collectivité territoriale à part entière et à fiscalité propre. » Le rapport de la Cour des comptes ne tarit pas d'éloges sur le bien-fondé de l'intercommunalité et sur ses bénéfices pour la solidarité territoriale, grâce à ses outils de créativité et d'inventivité.

tarifs de l'énergie incontrôlables ; fermeture d'écoles et de services ; factures de transfert d'enfants résidents vers d'autres communes à plus de 2 400 euros par enfant ; chats et chiens errants ; incivilités, etc.

en subissent toutes les nuisances. La France compte 34 950 communes et 1 250 EPCI. Ma question est simple, madame la ministre : que prévoyez-vous, rapidement et à terme, pour le devenir des maires et des communes françaises ? La parole

Plus globalement, vous vous interrogez sur la place et le rôle des communes et des EPCI dans notre organisation institutionnelle et territoriale. Sur le premier point, je rappellerai simplement les propos qu'a tenus Christophe Béchu au Sénat lors de son audition devant la commission des lois le 9 novembre 2022 : « J'ai lu le rapport de la Cour des comptes, je dois vous dire mon hostilité totale à l'idée que l'on pourrait transférer la DGF aux intercommunalités. [ ...] Remonter toute la DGF à l'intercommunalité, ce serait créer un dispositif qui créerait un remède pire que le mal. J'y suis donc totalement opposé. » Je vous le confirme : traduite, madame la sénatrice, dans la loi de finances pour 2023 récemment adoptée, qui a abondé la DGF des communes de 320 millions d'euros, dont 200 millions d'euros pour les communes les plus rurales et les plus fragiles.

Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place, au moment de la crise de la covid-19, puis de la poussée inflationniste, différents filets de sécurité et dispositifs de soutien, largement discutés et amendés par les parlementaires, afin d'aider les collectivités, notamment celles dont les ressources sont les plus contraintes, à traverser cette période si complexe. Nous ne mettons absolument pas en opposition frontale les communes et les EPCI. Au contraire, nous avons fait le choix de les accompagner en un même mouvement. Au-delà de cas particuliers problématiques, l'intercommunalité a

L'intercommunalité est un formidable instrument lorsque les élus communaux qui en assurent la gouvernance recherchent le consensus et s'accordent pour mettre en place les outils de solidarité territoriale qui, en vertu du principe de libre administration, sont à leur entière disposition.

Nombre de communes sont confrontées sur ces zones à des installations sauvages, souvent réalisées au vu et au su des autorités. Les auteurs des infractions se savent, la plupart du temps, à l'abri des poursuites et des sanctions du fait des contraintes légales et budgétaires qui pèsent sur les collectivités pour faire constater et cesser ces infractions. La loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a mis en place un nouveau mécanisme administratif de traitement des infractions aux règles d'urbanisme qui complète fort utilement les poursuites pénales. Je tiens à le souligner. heurte, dans la réalité, à de multiples obstacles de mise en oeuvre, qui vont de la difficulté de faire constater l'infraction face à l'hostilité des occupants illégaux jusqu'à l'impossibilité de faire recouvrer le montant des astreintes, ces mêmes occupants ayant bien souvent organisé leur insolvabilité. Certaines communes pensaient avoir trouvé la parade en préemptant, quand c'était financièrement faisable, des terrains sensibles lorsqu'une vente était annoncée. Mais désormais, ces terrains sont loués avec un bail emphytéotique, qui qui n'est pas soumis à la publicité foncière. La transaction passe ainsi sous les radars. À l'heure du « zéro artificialisation nette » (ZAN), la colère des élus locaux face à ces installations sauvages est compréhensible. Ils demandent que des moyens renforcés soient attribués à la justice et à la police de l'environnement, pour que ces dossiers soient traités rapidement, notamment dans les cas de mise en danger des personnes et de destruction de zones naturelles et agricoles. Les délais de procédure sont tels aujourd'hui qu'un dossier pour déboisement illégal, par exemple, ne sera toujours pas jugé quand le terrain sera totalement remblayé, viabilisé, construit et habité. Les dommages sont souvent irréversibles, et une fois un terrain habité, il sera pratiquement impossible de déloger un foyer installé. Aussi, madame la ministre, comment entendez-vous venir en appui des collectivités, pour que ce problème majeur soit traité efficacement et pour que la loi soit respectée dans sa plénitude ? La parole

en déterminant les secteurs dans lesquels les constructions sont interdites, ils permettent de mieux identifier les constructions illégales et en facilitent,, la verbalisation. La surveillance foncière des secteurs, notamment les plus sensibles d'entre eux, qui sont propices à des implantations discrètes et illégales, peut s'opérer dans le cadre des déclarations d'intention d'aliéner transmises aux communes en cas de vente de terrains et qui permettent de repérer les transactions atypiques pouvant donner lieu à des implantations illégales. Toutefois, comme vous l'avez relevé, la tâche est rendue plus difficile lorsqu'il y a non pas une cession préalable

le raccordement étant interdit pour les constructions illégales. Les infractions relevées pourront ensuite être traitées dans le cadre des procédures pénales, un outil qui ne doit pas être négligé. Certes, leur efficacité dépend de l'intervention effective de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, mais des protocoles de travail existent entre les services déconcentrés de l'État et les parquets, afin d'accompagner techniquement les maires. La loi du 27 décembre 2019 que vous mentionnez a instauré un mécanisme administratif rapide, qui est à la main des élus locaux parallèle aux poursuites pénales. Il permet la mise en demeure de régulariser, sous astreinte, les constructions, travaux et installations réalisés illégalement, y compris en cas de démolition nécessaire. Certes, comme vous l'indiquez, l'astreinte perd de son efficacité en cas d'insolvabilité de l'intéressé. Toutefois, elle peut viser non seulement le propriétaire, mais également toutes les autres personnes mentionnées par le procès-verbal d'infraction, comme les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou encore toute personne responsable de l'exécution desdits travaux. Le nombre élevé des personnes pouvant être visées par cette astreinte participe grandement à l'efficacité de l'outil. Il faut enfin rappeler que les services locaux de l'État peuvent assister les communes dans la lutte contre ces infractions, de manière directe ou au travers des divers guides élaborés à cette fin. En résumé, si le problème que pose la lutte contre les constructions illégales est prégnant,

Difficultés pour trouver un médecin traitant, retards de prise en charge, renoncements à des soins, allongements des délais d'attente : voilà ce qu'observent chaque jour les collectivités dont le territoire est frappé par la désertification médicale. Elles sont en première ligne face aux problèmes que rencontrent leurs habitants dans l'accès aux soins. En dépit des moyens limités dont elles disposent en matière de santé, elles sont nombreuses à prendre des initiatives,

d'information. Certains territoires proactifs mènent ainsi des politiques incitatives, afin de favoriser l'installation de médecins généralistes et spécialistes. Certaines collectivités proposent par exemple aux étudiants en médecine venus réaliser un stage sur leur territoire le versement d'indemnités d'hébergement et de transport. Leur action semble toutefois limitée par les dispositions de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales,

en ne s'adressant qu'aux étudiants de troisième cycle, le code général des collectivités territoriales ignore la réalité du parcours de ces étudiants qui, bien avant d'entamer leur troisième cycle, doivent déjà réaliser des stages. Madame la ministre, alors que ces aides constituent un levier efficace pour aider les collectivités à attirer de jeunes médecins, le Gouvernement est-il prêt à renforcer les compétences des collectivités en la matière et, plus précisément, à élargir

consistant en l'octroi d'aides à l'investissement ou au fonctionnement à tous les professionnels de santé, et elles peuvent verser une indemnité d'étude et de projet professionnel, ainsi qu'une indemnité de logement et de déplacement, aux stagiaires. Pour accompagner les étudiants, vous proposez d'étendre le bénéfice des indemnités de logement et de déplacement, actuellement limitées aux étudiants de troisième cycle de médecine générale, à l'ensemble des étudiants de médecine. Concernant l'extension du bénéfice de ces indemnités aux étudiants inscrits en troisième cycle de médecine spécialisée, le Gouvernement est favorable à cette proposition. En effet, les habitants des zones sous-denses rencontrent également des difficultés d'accès à la médecine spécialisée. Par ailleurs, une telle proposition est cohérente avec l'économie générale du dispositif prévu à l'article L. les indemnités d'étude et de projet professionnel peuvent d'ores et déjà être octroyées aux futurs médecins spécialistes. En revanche, étendre le bénéfice de ces indemnités à tous les étudiants en médecine, quel que soit leur cycle d'études, ne nous paraît pas répondre à votre objectif. En effet, ces indemnités ont vocation à prendre en charge les coûts liés à la réalisation d'un stage long de pratique professionnelle sur le territoire de la collectivité et à les sensibiliser à la pratique en zone sous-dense sans obligation d'installation ultérieure. Accompagnant la formation académique, les stages de premier et de deuxième cycle sont principalement réalisés dans des centres hospitaliers universitaires, qui sont situés dans des zones urbaines, et très peu dans des cabinets ou maisons de santé situés en zone sous-dense. La proposition ne nous paraît donc pas de nature à favoriser l'installation de jeunes médecins en zone sous-dense, contrairement aux indemnités d'étude et de projet professionnel, qui financent une formation dans son ensemble en contrepartie d'une obligation d'installation pendant au moins cinq ans, garantie par contrat. Enfin, je précise que le Gouvernement réfléchit à une extension du bénéfice

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, promise par le Président de la République lors de sa visite dans le département de l'Aisne en novembre 2018 dans le cadre de la signature du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache, la mise à 2x2 voies de la RN2 met un terme à quarante ans d'atermoiements sur ce dossier que tous les acteurs du territoire croyaient enlisé. Les objectifs du projet sont nombreux : désenclaver le nord de l'Aisne, réduire l'importante accidentalité de certaines portions de route et faciliter les connexions sur cet axe majeur qui relie le bassin parisien à la Belgique. Néanmoins, selon la décision ministérielle du 8 novembre 2022, la portion reliant Marle à Avesnes-sur-Helpe bénéficiera non pas du classement en route express à 110 kilomètres par heure, mais plutôt d'un aménagement en 2x2 voies à 90 kilomètres par heure. Cette décision déconcerte les acteurs économiques, ainsi que les élus du territoire. La patience dont ils ont su faire preuve pendant des décennies dans l'attente de cet équipement structurant ne semble pas être récompensée à sa juste valeur, mais se voit plutôt plutôt rétribuée par une proposition au rabais de la part de l'État. On peut bien évidemment entendre et comprendre les raisons liées au respect du paysage bocager de la Thiérache au nord de Vervins. Mais il apparaît tout à fait justifié de prolonger le classement en route express sur l'axe entre Marle et Vervins, qui traverse une importante zone d'activité économique et qu'il convient donc d'irriguer convenablement. Il est primordial que la concertation se poursuive sur les dernières modalités du projet. Madame la ministre, dans quel délai la déclaration d'utilité publique pourra-t-elle être publiée en vue de la poursuite des travaux ? Par ailleurs, quelle réponse entendez-vous apporter aux partisans d'une extension en voie rapide de la portion de RN2 destinée à

par décision du 8 novembre 2022, le ministre chargé des transports a retenu le principe d'un aménagement de la RN2 homogène à 2x2 voies sur l'ensemble du tronçon entre Laon et Avesnes-sur-Helpe. Cette décision confirme l'engagement de l'État pour ce territoire, en cohérence avec le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache que vous avez mentionné. Concernant le statut de route express, il convient de rappeler que ce statut implique de nombreuses contraintes, notamment en matière d'artificialisation des sols et d'émissions de CO2. Afin de concilier au mieux les enjeux de développement du territoire et ceux qui sont relatifs à l'activité agricole et à l'insertion environnementale, et en accord avec les conclusions de la concertation publique tenue en 2022, la décision ministérielle retient, sur cette différenciée en fonction des tronçons. L'aménagement de la RN2 entre Marle et Vervins se fera déjà en grande partie en tracé neuf, avec le contournement de trois communes, et sera consommateur d'emprises agricoles. Le choix d'un statut de route express sur la section entraînerait un impact foncier encore plus important résultant de l'aménagement complémentaire de voies de substitution pour les engins agricoles interdits sur route express. Les trafics sur cette section sont parmi les plus faibles de l'itinéraire- moins de 5 000 véhicules par jour en 2019. Les contraintes environnementales sont plus fortes qu'au sud de Marle, le tracé longeant notamment deux rivières. Au vu des impacts supplémentaires sur l'environnement et les activités agricoles, le faible gain de temps supplémentaire d'un aménagement à 110 kilomètres par heure avec statut de route express ne paraît pas justifier ce dernier sur une telle section. Pour l'avenir, les études vont se poursuivre sur l'ensemble de l'itinéraire, dont la section comprise entre Marle et Vervins, pour définir les variantes de tracés et proposer une analyse comparative qui fera l'objet de nouvelles concertations avec le public, avant de pouvoir présenter la variante retenue en enquête préalable

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les Ardennes sont affectées par de trop nombreux accidents ferroviaires, dont le dernier a été- hélas ! -mortel. À Donchery, c'est un père de famille et sa fille qui ont été percutés par un train de marchandises. L'enquête pour homicide involontaire n'a pas encore abouti, mais les faits sont malgré tout troublants, et même inquiétants, pour notre réseau : un système de signalisation défaillant ; une passerelle pour piétons datant des années 1940, vétuste et non utilisée- il n'y a donc pas d'autre choix que de traverser les voies un maire qui alerte en vain sur cette situation depuis des années et qui réclame des aménagements. Cet accident tragique illustre les problèmes que nous connaissons dans l'entretien des structures ferroviaires et de la signalisation.

En guise de réponse, la SNCF se défausse sur nos communes, qui n'ont ni les moyens ni les compétences pour assurer cette sécurisation. Les maires n'osent même plus demander des moyens par peur de voir une gare supprimée ... Voilà où nous en sommes en France en 2023 En 2013, à la suite de l'accident de Brétigny-sur-Orge, un plan d'action, Vigirail, avait été mis en place pour assurer la maintenance des voies et un niveau de sécurité renforcé. Où en est-on ? pas à surfer sur un drame humain, mais le nombre des récurrences frappantes m'autorise à vous dire que rien ne va plus ! Qu'envisagez-vous pour qu'il soit mis fin à ces défaillances ? À quelle fréquence les visites de contrôle sont-elles effectuées ? J'attends votre aide, madame la ministre, pour mettre la pression sur la SNCF, afin qu'elle daigne faire les travaux attendus depuis des années. N'attendons pas un drame supplémentaire Madame la ministre, vous

S'agissant plus spécifiquement des passages à niveau, les accidents ou collisions sur ces passages sont rares, mais souvent très graves. L'État s'est engagé en 2019 dans un plan d'action ambitieux pour améliorer leur sécurisation. sécurisation. Malheureusement, la sécurité aux passages à niveau relève aussi, voire principalement, de la sécurité routière : environ 98 % des accidents aux passages à niveau sont dus à des comportements à risque des usagers de la route. Les circonstances de chaque accident sont spécifiques. Les enquêtes ouvertes sur les événements que vous évoquez permettront d'en déterminer les causes. En tout cas, je veux réaffirmer devant vous l'engagement du Gouvernement de ne pas transiger sur l'effort de remise à niveau et de modernisation de notre réseau ferroviaire. Le contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau y consacre un niveau de dépenses historiquement élevé. Nous irons plus loin, en lien avec les préconisations du Conseil d'orientation des infrastructures. La parole

à la fin du mois de novembre dernier, la SNCF décidait unilatéralement de nouvelles modifications d'horaires sur la ligne Intercités Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, dite Polt, entraînant une absence totale de liaison entre l'ancienne région Limousin et la capitale une partie de la matinée, avec toutes les conséquences économiques et sociales que cela représente pour les entreprises locales et les usagers.

Depuis trente ans, tel est le quotidien des habitants qui utilisent cette ligne : modifications d'horaires et suppressions de trains sans solutions de substitution fournies par la SNCF ; retards systématiques atteignant parfois plusieurs heures ; accidents à répétition. La situation est tellement critique que le groupe Legrand- l'une des seules entreprises du CAC 40 ayant son siège en province -a clairement évoqué un risque de départ. Le porcelainier Bernardaud a fait état de sérieuses difficultés dans son développement et de nombreuses entreprises signalent des pertes de chiffre d'affaires du fait de ces difficultés d'accès. notamment en charge de la ruralité : êtes-vous prête à assumer une telle catastrophe pour notre territoire ? À court terme, la SNCF s'est engagée, entre autres, sur l'amélioration significative du fonctionnement des trains durant l'hiver et sur l'arrêt des suppressions d'horaires. Mais les usagers de cette ligne attendent davantage : le rétablissement des quatorze allers-retours qui existaient jusqu'en 2015, avec desserte des gares intermédiaires, ainsi que le développement du fret et des trains de nuit. Pouvez-vous m'assurer que les délais annoncés pour les travaux de régénération de la ligne et la livraison des nouvelles rames seront tenus et que la modernisation qui mettrait Limoges à deux heures trente de la capitale sera engagée, avec en particulier la commande de rames supplémentaires, seul moyen sérieux d'y parvenir ?

je partage votre constat. En ce qui concerne le déraillement d'un train de fret en décembre à Issoudun, je souhaite tout d'abord rappeler que l'enquête est toujours en cours pour en déterminer les responsabilités. Je remercie par ailleurs la SNCF du travail effectué pour relever ce train dans des conditions difficiles. La réduction du plan de transport cet hiver sur la ligne Paris-Limoges-Toulouse est largement due au faible nombre de locomotives racleuses mises à disposition par SNCF Réseau pour traiter le givre, et cela malgré une amélioration partielle de la situation grâce à la mise en service par SNCF Intercités, à ses propres frais, d'une locomotive racleuse supplémentaire. Le ministre chargé des transports a clairement exprimé son exigence au gestionnaire d'infrastructure, qui devra revoir son parc de locomotives racleuses dès l'hiver prochain, dans l'attente des nouvelles rames Oxygène qui circuleront dès 2025 sur la ligne et qui pourront être équipées de pantographes racleurs. Au-delà de ces problèmes saisonniers, le Gouvernement a demandé au groupe SNCF des actions concrètes pour améliorer la qualité de service sur cette ligne primordiale pour assurer convenablement la desserte de nos territoires. À cet effet, un groupe de travail technique réunira trimestriellement l'État, le groupe SNCF et le monde économique et associatif, ainsi que les parlementaires et les élus du territoire, pour rendre compte de la mise en oeuvre de ce plan d'action et évaluer l'amélioration de la qualité de service. Le ministre chargé des transports participera à la première réunion de ce groupe de travail technique à Limoges à la fin du mois de février prochain.

dix départements traversés, et une vingtaine qui lui sont reliés. Cette ligne structure directement la vie économique et touristique de ce territoire, en assurant la liaison entre Paris et la province. Mais encore faut-il que les trains roulent ! Le

Urgence Ligne Polt pour défendre cette ligne. Au cours des trente dernières années, cette ligne a malheureusement été délaissée pendant qu'un TGV hypothétique- et non financé ! -était envisagé entre Limoges et Poitiers.

De plus, il faut absolument que le plan de régénération de 400 millions d'euros destiné à réduire le temps de trajet d'un quart d'heure soit réalisé. Madame la ministre, vous êtes garante de l'égale répartition des chances entre les territoires de notre République une et indivisible. Comment l'État s'assure-t-il que la SNCF mette bien à disposition de la ligne Polt les ressources humaines et matérielles nécessaires au retour d'un service de qualité en toutes circonstances ?

Cette ligne va bénéficier d'investissements significatifs de la part de l'État : l'arrivée d'un nouveau matériel roulant, dont le financement s'élève à 450 millions d'euros, et un programme de modernisation visant à améliorer les performances de la ligne d'ici à 2026, dont les deux tiers seront financés par l'État, à hauteur de 257 millions d'euros, le tiers restant ayant vocation à être apporté par les régions concernées et intéressées par l'amélioration de la performance de la ligne. Par ailleurs, des travaux de régénération entièrement financés par SNCF Réseau sont réalisés jusqu'en 2025, afin de remettre à niveau l'infrastructure pour un montant total de 1,6 milliard d'euros.

Pour l'hiver 2022-2023, SNCF Réseau a augmenté de 50 % le nombre de trains racleurs déployés. Les autres techniques de dégivrage mobilisées sont le réchauffage de la caténaire ou encore le décalage des circulations pour éviter la reformation de givre. Afin d'assurer un suivi plus régulier associant les parties prenantes, le ministre chargé des transports a demandé à la SNCF la mise en place d'un groupe de travail technique se réunissant à fréquence trimestrielle et se concentrant sur les améliorations de la qualité de service. Je vous confirme ainsi l'engagement du Gouvernement pour l'amélioration de la robustesse et de la qualité de service de la ligne Polt

en se fondant sur l'existence de cette ligne et sur sa pérennité. Sa fermeture définitive ne peut donc pas être acceptée par les chefs d'entreprise qui ont fait le choix d'implanter leurs activités sur le territoire du fait des facilités économiques qu'elle

enregistrait en 2019 un taux d'occupation de moins d'un siège sur trois et accusait chaque année un déficit particulièrement élevé. Cette liaison a été suspendue en 2020 en raison de la crise sanitaire. Depuis la fin de celle-ci, la tendance structurelle de baisse du trafic professionnel et du trafic en correspondance depuis l'aéroport de Roissy a encore accentué le déséquilibre financier. SNCF Voyageurs est conscient des difficultés que cela peut poser aux clients qui préféraient une liaison directe, mais l'entreprise doit chercher à concilier les objectifs de gains de performance et de contribution au développement des territoires. Néanmoins, des échanges Néanmoins, des échanges ont déjà été engagés par SNCF Voyageurs avec les acteurs locaux sur le sujet. À la suite de cette concertation, l'offre de service du dimanche entre Paris et Montbard s'est enrichie d'un aller-retour depuis le 11 décembre 2022, ce qui a d'ailleurs été salué par les acteurs du territoire. Il faut aussi rappeler que l'offre entre Paris et Montbard, dont la fréquentation est pourtant en baisse du fait des évolutions liées au télétravail, restera inchangée en semaine en 2023, avec quatre allers-retours quotidiens. Enfin, la qualité de l'offre de la Bourgogne depuis et vers Paris, en particulier pour Dijon, qui dispose d'une desserte dense, permet de proposer plusieurs possibilités en correspondance. Les échanges se poursuivent en vue d'identifier une solution qui puisse concilier les attentes de l'ensemble des parties prenantes ; ces discussions sont en bonne voie.

Certaines collectivités ne sont plus en mesure de compenser le différentiel entre les montants initiaux et ceux qui sont actualisés. Vous savez, madame la ministre, que ces projets sont parfois vitaux pour les petites communes et nos territoires ruraux. C'est par exemple le cas d'un projet de requalification de centre-bourg dans la commune d'Orgueil, dans mon département, le Tarn-et-Garonne. Sur un projet d'environ 820 000 euros, la commune avait obtenu 640 000 euros de financement, avec un reste à charge de 180 000 euros. Compte tenu de la crise de l'inflation et de la nécessité de relancer le marché initial déclaré infructueux, le surcoût des travaux s'est élevé à 44 % et le reste à charge pour la commune est finalement de 480 000 euros : 300 000 euros de plus que le montant initial, ce n'est pas tenable pour le budget de cette petite commune En l'état, la commune d'Orgueil, comme des milliers d'autres qui sont dans le même cas, devra certainement renoncer à ses projets stratégiques. En parallèle, la préfecture du Tarn-et-Garonne aurait, en 2022, rendu 1 million d'euros de DETR non consommée au titre des années précédentes. Ne serait-il pas possible de redéployer les crédits annuels non consommés sur l'appel à projets suivant, dans une dotation complémentaire destinée aux dossiers subissant d'importants surcoûts ? Ou ne serait-il pas envisageable de prendre en compte les surcoûts générés par l'inflation, en faisant entrer celle-ci dans la part subventionnable de la DETR et de la DSIL lorsque cette part n'est pas à son maximum ? De façon plus générale, madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer les moyens que vous comptez mettre en oeuvre afin de soutenir l'investissement local dans un contexte de forte inflation ? Je vous remercie par avance de votre réponse, qui sera scrutée par des milliers de maires et de présidents d'intercommunalités. La parole

avec près de 2 milliards d'euros en autorisations d'engagement- et même 4 milliards d'euros en incluant le fonds vert -, le soutien de l'État à l'investissement local est maintenu à un niveau particulièrement élevé, afin d'accompagner au mieux le dynamisme des territoires. Vous avez raison, dans un contexte d'inflation, les collectivités peuvent faire face à davantage de difficultés dans le financement des projets d'investissement qu'elles souhaitent porter. L'État les accompagne dans ces projets, en apportant un soutien financier qui peut aller jusqu'à 80 % des financements publics. ajoutée (FCTVA), qui intervient en moyenne à hauteur de 16 %, et ce sur la base du montant définitif des dépenses éligibles. En principe, il n'est pas possible d'augmenter le taux de subvention DETR ou DSIL figurant dans l'arrêté attributif. Il s'agit d'une règle de bonne gestion budgétaire, permettant de sécuriser la trajectoire des dépenses. Cela inclut le cas où un projet, déjà subventionné, connaîtrait en cours de réalisation des surcoûts par rapport aux montants initialement prévus par les communes et intercommunalités. Il est néanmoins envisageable, si les projets peuvent être scindés en plusieurs tranches distinctes, d'octroyer une nouvelle subvention correspondant à une nouvelle tranche ne portant pas sur la même assiette. Il est également possible de solliciter un autre levier de financement pour compenser au mieux cette augmentation du coût à l'aide par exemple de la DSIL pour un projet subventionné par la DETR, et inversement, les deux dotations étant cumulables. En dernier lieu, le droit de dérogation du préfet, prévu par le décret du 8 avril 2020, permet également, sous certaines conditions, de modifier le taux de la subvention attribuée. Il convient toutefois de l'employer à bon escient pour que cette règle budgétaire ne perde pas sa portée. Il convient en particulier de s'assurer qu'il existe un risque réel d'abandon du projet, et ce malgré l'absorption par le titulaire du marché d'une part de la hausse du coût. En effet, la puissance publique- collectivités et État -ne doit pas supporter seule l'intégralité de la hausse des prix. En ce qui concerne le redéploiement des crédits que vous proposez, dans les faits, la quasi-totalité des crédits mis à disposition des préfectures est effectivement consommée chaque année. Le principe d'annualité budgétaire prévu par la loi implique que les crédits soient ouverts uniquement pour l'année en cours. Il impose ce faisant un haut niveau de consommation. Il a également pour conséquence que les redéploiements entre opérations ne peuvent se faire qu'au sein d'un même exercice annuel. Les montants tout à fait résiduels- quelques dizaines de milliers d'euros sur plus de 2 milliards d'euros en autorisations d'engagement -qui n'ont pas pu être consommés pour des raisons techniques sont reportés en totalité sur l'exercice suivant.

conserve encore aujourd'hui un rôle majeur. Il a résisté aux crues successives, dont celles de 2002 et 2003, qui restent dans toutes les mémoires des Caderoussiens et, plus largement, des Vauclusiens. Il est d'ailleurs classé « ouvrage intéressant la sécurité publique » par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2006.

des herbes et arbustes dans les joints. En effet, depuis le 1 juillet 2022, l'utilisation des produits phytosanitaires pour détruire les végétaux qui se développent entre les pierres est interdite aux personnes publiques, et

des modalités alternatives » pour désherber les talus par des moyens thermiques, mécaniques ou de biocontrôle. Madame la ministre, le maire de Caderousse et moi-même sommes bien conscients des enjeux écologiques et et comprenons que l'utilisation de ces produits phytosanitaires doit être raisonnée et limitée dans le temps et dans l'espace. Cependant, aujourd'hui, les produits de biocontrôle proposés ne permettent pas de contenir efficacement les racines des végétaux. Il existe des dérogations à l'interdiction des produits proscrits, par exemple lorsqu'un danger sanitaire grave vient à mettre en péril la pérennité du patrimoine historique. Ne pensez-vous pas, madame la ministre, que le risque d'inondation, avec ses enjeux humains, économiques et environnementaux, constitue un danger grave qui pourrait justifier la mise en place d'une telle dérogation ? La parole est à Mme la ministre déléguée.

Labbé de 2014 interdisant l'usage des produits phytosanitaires dans les espaces verts publics. En effet, il souhaite pouvoir désherber avec des pesticides conventionnels les digues d'enceintes de la ville, qui datent de 1856 et qui sont classées au titre des monuments historiques. Tout d'abord, je rappelle que l'utilisation des produits phytosanitaires est interdite depuis le 1 janvier 2017 pour l'entretien des espaces verts, des voiries ou des promenades accessibles au public. Le maire de Caderousse a demandé en 2022 au directeur

biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique. Il convient d'examiner la possibilité d'utiliser dans ce cas, comme le font déjà de très nombreux maires, des moyens thermiques ou mécaniques pour éradiquer les mauvaises herbes et les plants d'arbustes. La technique du brûlage se révèle ainsi efficace pour pour lutter contre le maintien des racines dans les interstices des pierres. J'ai demandé au directeur de l'eau et de la biodiversité d'examiner les conditions dans lesquelles le plan Écophyto pourrait être mobilisé pour soutenir le traitement de tout ou partie des remparts de la ville. Je vous invite à prendre contact avec les équipes du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires pour déterminer les conditions précises d'un tel soutien. La parole est

d'eau potable sont perdus chaque année, ce qui représente l'équivalent de 300 000 piscines olympiques. Alors que nous faisons face à des sécheresses de plus en plus importantes, nous devons plus que jamais préserver cette ressource. Sans eau, point de vie ! Il est donc indispensable de donner à nos collectivités locales les moyens de mettre en oeuvre les travaux nécessaires pour remédier à la vétusté du réseau. En effet, en certains endroits, il y a de véritables passoires, à cause du vieillissement des canalisations, de la corrosion, des glissements de terrain ou d'autres avaries. En Gironde, dans la commune de Langoiran, les chiffres révélés par le syndicat des eaux font apparaître un indice linéaire de perte de 7 200 litres d'eau par kilomètre chaque jour-

Dans le Blayais, la déperdition en eau potable est également considérable. Le syndicat des eaux a cependant entrepris des travaux pour renouveler les canalisations, notamment celles en fonte, qui sont la cause des eaux rouges, pour un coût de plus de 1,5 million d'euros entre 2022 et 2023. Bien que le décret potable impose aux collectivités d'atteindre un certain seuil de rendement pour leur réseau, les travaux nécessaires représentent un coût rédhibitoire. Sans un accompagnement financier de l'État, il sera difficile pour nos communes de les mettre en oeuvre. Or ils sont essentiels d'un point de vue environnemental.

le premier chantier de planification de la préservation de la ressource en eau. La concertation qui s'est ouverte a mobilisé l'ensemble des comités de bassin, le Comité national de l'eau, ainsi que les collectivités. Elle va aboutir rapidement à un plan eau, qui fixera une ambition politique commune, autour, notamment, des enjeux que vous mentionnez. Dans le cadre du plan de relance, les agences de l'eau ont engagé en 2021 près de 250 millions près de 250 millions d'euros d'aides pour des projets portant sur la modernisation du réseau d'eau potable, la mise aux normes de stations de traitement des eaux usées, la rénovation des réseaux d'assainissement, le déraccordement des rejets d'eaux pluviales et leur infiltration à la source, ainsi que sur l'hygiénisation des boues d'épuration. Ces crédits sont venus renforcer les moyens mis en oeuvre au titre des onzièmes programmes d'intervention des agences, qui prévoient 4,5 milliards d'euros d'aides sur le petit cycle de l'eau, dans la lignée des engagements pris lors des Assises de l'eau, notamment en faveur des collectivités en zone rurale. ailleurs, un premier relèvement du plafond de dépenses des agences de l'eau en 2022, complété par un second en 2023, chacun à hauteur de 100 millions d'euros, a accru les possibilités d'appui aux collectivités sur ces sujets. particulièrement vocation à accompagner les investissements des collectivités qui ont été confrontées à une rupture ou un risque de rupture d'approvisionnement en eau potable l'été dernier. Les agences de l'eau et l'Office français de la biodiversité vont enfin faire porter leur effort plus spécifiquement sur la lutte contre les fuites d'eau, grâce à une dotation de 50 millions d'euros accordée dans la loi de finances rectificative pour 2022. ciblées sur les territoires les plus fragiles ou sur les situations les plus critiques, viennent compléter l'offre de prêts de la Banque des territoires, dite Aqua Prêt, dont le taux compétitif et l'échéance, adaptée à la durée d'amortissement des investissements, devraient permettre d'accompagner l'ensemble des services publics publics d'eau et d'assainissement dans leurs travaux. Concernant le Syndicat des eaux du Blayais, l'agence de l'eau Adour-Garonne a accordé en 2016 et 2020 des aides pour le renouvellement des réseaux d'eau potable, pour un montant de 615 000 euros.

Madame la ministre, je souhaite vous interroger sur l'obligation faite au policier municipal qui serait également sapeur-pompier volontaire de déposer son arme dans le coffre du poste de police dans lequel il exerce. C'est le maire de Cazouls-lès-Béziers, dans l'Hérault, qui m'a interpellé à sujet. Face à la pénurie de sapeurs-pompiers volontaires, les policiers municipaux ont intégré les centres de secours afin de renforcer les effectifs, surtout en journée, ce qui est une bonne chose. Cependant, comme toujours, le diable se cache dans les détails,

pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l'arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité.

vous avez interrogé M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérard Darmanin, qui, ne pouvant être présent, m'a chargée de vous répondre. L'article 114-4 du règlement issu de l'arrêté du 6 juin 2006 que vous mentionnez concerne les policiers nationaux et n'est donc pas applicable aux policiers municipaux. C'est l'article R. 511-32 du code de la sécurité intérieure qui fixe les conditions de dépose des armes des policiers municipaux. Cet article dispose que, sauf lorsqu'elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation [ ...], les armes [ ...] et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte scellés au mur et au sol d'une pièce sécurisée du poste de police municipale. » Le fait que ce policier municipal soit, par ailleurs, sapeur-pompier volontaire, n'est pas une raison suffisante pour le soustraire à cette obligation, qui s'applique à l'ensemble des policiers municipaux et constitue un gage de sécurité important. De surcroît, les casernes des services d'incendie et de secours ne sont pas conçues pour répondre aux mêmes exigences que les locaux de police municipale. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation en vigueur. La parole

de Canadairs. Le dérèglement climatique accentue les besoins en moyens visant à endiguer les départs et propagations de feux, notamment de feux de forêt, afin d'éviter la survenue de nouveaux mégafeux. Dans ce contexte, les Canadairs sont un outil indispensable. À ce titre, le 7 mai 2020, la direction générale de la sécurité civile a transmis une demande à la direction générale de l'armement (DGA) pour le lancement du marché d'acquisition de deux avions bombardiers d'eau amphibies. Ces deux appareils devaient être financés par le programme européen RescEU à 90 %, mais nous venons

La nouveauté de l'année 2022, c'est l'annonce par le Président de la République, le 28 octobre dernier, du renouvellement intégral de la flotte de Canadairs, qui doit en outre être renforcée pour passer de douze à seize appareils, dont les deux du programme RescEU, d'ici à la fin du quinquennat.

entre en contradiction avec les propos tenus par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi qu'avec les réponses fournies par la DGSCGC aux derniers questionnaires budgétaires. En effet, il était plutôt

précisiez les mesures que le Gouvernement entend mettre en place pour augmenter de manière substantielle les capacités de la flotte aérienne- groupement « avions » et groupement « hélicoptères » -, dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt. Mes chers

des douze Canadairs est un outil indispensable et particulièrement efficace. Elle est augmentée par la participation de la France au mécanisme de protection civile de l'Union européenne (MPCU) et au programme visant la création d'une réserve de sécurité civile européenne (RescEU). À terme, douze avions

Dans cette perspective, la DGSCGC a officiellement fait une demande à la DGA pour acquérir deux avions amphibies bombardiers d'eau le 7 mai 2020, sur la base d'un cofinancement validé par la Commission européenne le 18 novembre 2020. Le marché considéré prévoit la possibilité de commander deux avions supplémentaires sur fonds propres de la DGSCGC, ce qui porterait ainsi à seize le nombre d'avions amphibies bombardiers d'eau. De plus, le Président de la République a annoncé, le 28 octobre dernier, non seulement la modernisation de notre flotte de Canadairs, mais également l'acquisition de quatre aéronefs supplémentaires pour porter à Concernant le point très spécifique du retard pris par la société Viking Air, devenue De Havilland Canada, un dialogue a été engagé depuis de nombreux mois entre la société, la Commission européenne et les États membres. Ces échanges ont abouti le 31 mars dernier à un déblocage du projet et à une officialisation du lancement de la chaîne de production des nouveaux avions amphibies bombardiers d'eau, avec cependant un glissement du du calendrier de livraison, qui reste encore à déterminer. En outre, la France dispose de trois Beechcraft pour la phase de reconnaissance et de coordination, ainsi que d'une flotte d'avions Dash en charge des missions de guet aérien armé et de l'attaque des feux naissants, avec la pose de barrières de retardant. Le huitième et denier appareil de la flotte sera livré au premier semestre 2023. Par ailleurs, des discussions sont engagées avec la Commission européenne

Son cas n'est malheureusement pas isolé. Je dois vous dire que cette mésaventure m'est également arrivée, et plusieurs autres personnes se trouveraient dans cette situation, que l'on peut qualifier de troublante, voire d'absurde. Dans un article paru dans la presse en décembre 2020, le préfet de la Sarthe expliquait que, pour le renouvellement de leurs pièces d'identité,

être le mien : « J'ai vécu cette situation comme une humiliation, une insulte à ma famille, qui a été obligée de quitter l'Algérie, sa terre natale, en catastrophe, en laissant tout derrière elle. Une insulte à mon père, qui a combattu dans les rangs de l'armée française. »

Darmanin, qui, ne pouvant être présent, m'a chargée de vous répondre. Les rapatriés d'Algérie disposant de la nationalité française se voient en effet parfois demander la production d'un certificat de nationalité française ou se trouvent dans l'obligation de prouver leur nationalité à l'occasion du renouvellement de leur titre. Vous avez raison de le souligner, il a déjà été rappelé que, lors du renouvellement de leur carte nationale d'identité ou de leur passeport, les rapatriés d'Algérie n'ont pas à produire de certificat de nationalité française. En effet, une fois que la nationalité française est prouvée et que les documents d'identité à renouveler sont valides ou périmés depuis moins de cinq ans, les pièces du dossier demeurent dans le système titres électroniques sécurisés », et il n'est pas besoin de renouveler ces éléments. En revanche, lors du renouvellement d'un titre échu depuis plus de cinq ans, il est demandé de prouver sa nationalité. En effet, les éléments ne sont plus conservés dans le traitement de données, compte tenu des délais de conservation des données, et les anciens titres produits sont parfois contrefaits. N'importe quoi ! Aussi, s'il est constaté des manquements aux consignes de renouvellement simplifié des titres valides ou échus depuis moins de cinq ans, s'agissant des rapatriés d'Algérie disposant de la nationalité française, des instructions

J'attends encore des réponses concrètes. Madame la ministre, seuls 18 % de notre population occupent un emploi salarié. L'indice des prix à la consommation était de 4,6 % à la fin de 2022, et il continue d'augmenter. Le commerçant qui achète un conteneur d'eau minérale en France doit payer cinq fois plus pour le transporter vers notre territoire. Le coût du transport des marchandises conditionne les prix à la consommation, qui sont devenus incontrôlables, car ils dépendent des compagnies maritimes qui ont le monopole de la desserte. La population est également victime du laxisme des autorités, qui tolèrent, depuis 2017, depuis 2017, une taxe non réglementaire de 18 % appliquée par la chefferie coutumière sur toutes les marchandises, dont les produits de première nécessité. La seule banque de l'île, la BWF, contribue à asphyxier l'économie en bloquant l'activité des entreprises. Elle facture des frais exorbitants, refuse les ouvertures de compte, clôt abusivement les comptes privés et professionnels, et j'en passe ... Ce sont autant de freins pour notre développement économique. Madame la ministre, l'État est-il prêt à agir concrètement pour lutter contre la vie chère à Wallis-et-Futuna, d'une part, en créant un service de contrôle des prix pour garantir une pratique légale et cohérente et, d'autre part, en cofinançant l'achat d'un bateau qui sera exploité pour le territoire

Si l'inflation dans les îles de Wallis et Futuna est légèrement plus faible que dans l'Hexagone, elle s'applique à des prix initialement plus élevés. Pour faire face à cette situation, l'accord de modération des prix signé en 2022 comprend un bouclier qualité-prix regroupant 83 produits de grande consommation, soit 22 produits supplémentaires par rapport à celui de 2021. Il est en vigueur dans 18 points de vente. Cet accord et ces améliorations ont été rendus possibles par les efforts des opérateurs économiques, notamment du principal importateur grossiste du territoire, qui ont limité leur marge sur des produits de première nécessité. Le renforcement du bouclier qualité-prix constitue aussi un moyen de soutenir la production locale, puisque 14 produits locaux en font aujourd'hui partie. Nous souhaitons poursuivre ces efforts en nous inspirant de la démarche du « Oudinot du pouvoir d'achat », lancée dans les départements et régions de l'archipel à de nombreux secteurs et obtenir la contribution de nouveaux opérateurs, dont les acteurs du fret, qui ne sont pas aujourd'hui signataires de l'accord. En ce qui concerne le coût de l'énergie, Wallis-et-Futuna a intégré le dispositif national de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) et dispose à ce titre du bénéfice des tarifs réglementés

de la jeunesse. Madame la secrétaire d'État, vous le savez, la dimension territoriale des politiques publiques constitue la marque du Sénat. C'est pourquoi je souhaite vous interroger sur la déclinaison territoriale de l'enseignement scolaire en milieu rural. Les territoires français sont multiples et ils rencontrent des difficultés ou bénéficient d'avantages que nous devons examiner avec lucidité. C'est d'ailleurs grâce à ce constat objectif que les politiques de l'éducation nationale ont été pensées, puis ciblées. La définition de la carte de l'éducation prioritaire s'appuie ainsi principalement sur l'indice de position sociale (IPS), qui prend en compte les chances de réussite scolaire de l'élève à partir de la catégorie socioprofessionnelle de ses parents, de ses conditions matérielles de vie ou encore des pratiques culturelles dont il bénéficie.

Or, dans le monde rural, la part de la population pauvre ne se concentre pas dans un quartier prioritaire. La pauvreté est moins densément concentrée, mais elle y est tout aussi présente. La prise en compte de cette géographie sociale de notre pays est un impératif si l'on souhaite garantir le principe d'égalité entre les citoyens. Certes, il existe une politique d'allocation progressive des moyens pour les établissements écartés du réseau REP. Vous m'en avez déjà parlé dans cet hémicycle lors d'une précédente séance de questions orales. Cependant, nous sommes bien loin des moyens mis en oeuvre grâce au classement en REP le dédoublement des classes, la prime pour les personnels d'éducation, la formation spécifique, les moyens de coordination, etc. Madame la secrétaire d'État, je connais votre attachement à la justice sociale. Aussi, quand pensez-vous faire bénéficier ces écoles des secteurs ruraux éloignés et pauvres des mêmes moyens que l'éducation prioritaire des villes ? La

Les séjours éducatifs dans les centres d'hébergement, tels que les classes de neige ou les classes de découverte, contribuent à donner du sens aux apprentissages par le contact direct avec un nouvel environnement. Ils permettent aux élèves d'agir ensemble dans des situations et des lieux nouveaux.

Cette réalité de terrain affecte le développement de ces classes de découverte, pourtant essentielles à nos enfants, mais aussi au modèle économique de ces établissements et de certaines stations lors des « ailes de saison Avant la crise de la covid-19, une circulaire était en préparation pour simplifier cette procédure d'autorisation. À ce jour, elle n'est toujours pas parue. Madame la secrétaire d'État, le Gouvernement a-t-il prévu de simplifier cette procédure d'autorisation pour faciliter la mise en oeuvre des séjours éducatifs

En l'état, l'académie de Limoges devrait rendre 23 postes dans le premier degré et 18 dans le second degré. La Haute-Vienne est particulièrement touchée par ces suppressions de postes et fermetures de classes. Dans le premier degré, les chiffres sont évocateurs

Comment faire face au dédoublement des grandes sections ? Comment aller plus loin dans l'inclusion scolaire en supprimant des postes et en fermant des classes ? ne pensez-vous pas, madame la secrétaire d'État, qu'un moratoire sur la fermeture de classes s'impose ? Enfin, pourriez-vous m'expliquer comment la baisse des moyens humains pourrait permettre d'améliorer la qualité et la continuité du service public de l'éducation nationale, déjà fortement sous-doté en Haute-Vienne ? La parole

l'objectif de limiter le nombre d'indemnités journalières pouvant être touchées par une personne en situation de cumul emploi-retraite. Depuis lors, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) interprète de manière extensive ce dispositif, en l'appliquant aux personnes en situation de retraite progressive ne touchant qu'une fraction de pension. Depuis maintenant deux ans, nombre de ces retraités progressifs se sont retrouvés dans une situation intenable en cas d'arrêt maladie prolongé ou à répétition, touchant seulement une fraction de pension, mais plus de salaire, ni d'indemnité maladie. Dans certains cas, la CPAM a réclamé tardivement les indemnités indues à ces retraités progressifs, qui doivent ainsi rembourser des sommes considérables. La plupart de ces personnes ont dû prendre leur retraite de façon précipitée, y compris lorsqu'elles n'avaient pas tous leurs trimestres de cotisation, menaçant ainsi l'intérêt même du dispositif des retraites progressives, prévu pour faciliter l'emploi des seniors. Ma question est donc double : alors que le projet du Gouvernement est désormais de repousser l'âge de départ à la retraite, est-il prévu de modifier l'article L. 323-2 323-2 du code de la sécurité sociale pour en exclure les retraités progressifs ? Le cas échéant, cette modification pourrait-elle avoir un effet rétroactif, afin d'aider les personnes qui sont actuellement confrontées à cette interprétation injuste de la loi par la CPAM ?

aux assurés en retraite progressive, afin de ne pas pénaliser ces derniers, tout en favorisant les situations de maintien en activité des assurés en cumul emploi-retraite. Cette mesure s'inscrit dans l'objectif d'amélioration et de généralisation des dispositifs de transition entre l'activité et la retraite, afin de mieux préparer les fins de carrières, de favoriser des transitions douces et de permettre à ceux qui le souhaitent de travailler plus longtemps. Les améliorations du cumul emploi-retraite

2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer. En effet, cette loi a pour objet de rehausser à 85 % du Smic, soit 1 150 euros net par mois au 1 janvier 2023, la retraite minimum des anciens chefs d'exploitation agricole ayant eu une carrière complète. Cette revalorisation est entrée en application le 1novembre 2021, mais de nombreux

ce qui réduit d'autant et de manière significative la portée de la loi, dont l'application devient de ce fait assez lacunaire. De toute évidence, les bonifications pour enfants n'ont pas vocation à être prises en compte dans le calcul des pensions concernées. Que compte donc faire le Gouvernement pour

référence a vocation à porter les droits personnels de base et complémentaires servis par le régime de retraite des non-salariés agricoles à un montant minimal, tout en tenant compte des autres pensions personnelles de retraite perçues par l'assuré. Pour tenir compte de ces pensions, le complément différentiel fait l'objet d'un écrêtement. Autrement dit, si la somme de l'ensemble des pensions personnelles perçues par l'assuré et du complément différentiel calculé selon les dispositions de l'article D. 732-166-4

en particulier son deuxième alinéa, qui prévoit que les bonifications pour enfant afférentes aux pensions personnelles de l'assuré sont prises en compte pour l'écrêtement du complément. Le mouvement de revalorisation des petites pensions se poursuivra dans la réforme des retraites qui sera examinée au Parlement en ce début d'année 2023. La parole

la fonction publiques et concerne le cas des collectivités territoriales qui, faute de candidats à certains postes, ne peuvent pas satisfaire à leurs obligations légales.

sauf dispositions spécifiques prévues dans les statuts particuliers. Or de nombreuses collectivités territoriales peinent à recruter des agents pour des missions à horaires atypiques tels que les postes d'accompagnateurs de bus, qui ont pour rôle d'assister les enfants âgés de 3 ans à 6 ans utilisant les transports scolaires- une heure le matin et une heure l'après-midi, quatre jours par semaine.

je vous remercie

Depuis quelques années, les prises de rendez-vous pour une demande de visa sont externalisées à des prestataires privés, au lieu d'être effectuées par les postes consulaires dont les effectifs ne cessent de se réduire. Cette externalisation a eu des effets pervers, qui créent des inégalités de traitement inacceptables et nuisent fortement à l'image et à la réputation de notre pays. Tout d'abord, les demandes de visas des conjoints de ressortissants français, qui étaient auparavant gratuites, sont désormais soumises à des frais de prises en charge par le prestataire privé. Or les sommes sont parfois très importantes en rapport au niveau de vie local, notamment en Asie ou en Afrique. Pis encore, ces prestataires privés proposent des services additionnels facultatifs aux demandeurs de visa qu'ils vendent sous les dénominations trompeuses d'« offre premium » ou d'« offre VIP », à des prix exorbitants.

Enfin, l'externalisation de ces prises de rendez-vous a entraîné le développement d'officines, qui préemptent les créneaux de prise de rendez-vous auprès du prestataire pour les revendre à des prix abusifs. La pénurie de rendez-vous que ces officines provoquent à dessein laisse à penser aux demandeurs de visas qu'elles sont le seul recours pour obtenir un rendez-vous de dépôt d'un dossier de demande de visa.

partout où cela est possible, des dispositions sont prises pour faciliter leur accès aux services du prestataire, pour déposer une demande de visa. Dans une majorité de pays, des créneaux de rendez-vous sont clairement identifiés pour les demandeurs. Les conjoints de Français peuvent également déposer leur demande sans rendez-vous, sur simple présentation chez le prestataire d'un justificatif récent prouvant le lien matrimonial avec le ressortissant français. Enfin, si la règle veut que les demandeurs ne peuvent être accompagnés lorsqu'ils déposent leur demande de visa, les postes consulaires et les prestataires peuvent l'autoriser au cas par cas, en fonction du besoin exprimé et de la nécessité de l'accompagnement. Des consignes ont été passées, et même rappelées, pour qu'ils fassent preuve de souplesse s'agissant des conjoints de Français. Pour ce qui est des officines, et au-delà des rappels adressés à nos postes sur la gratuité de la prise de rendez-vous, plusieurs mesures de lutte

dire, car ce qui se passe est honteux. Ces mesures ont malheureusement parfois des effets limités, dans la mesure où le recours à une intermédiation pour les démarches administratives est très répandu dans certains pays,

Elle a donc subi un écrêtement de sa dotation forfaitaire conduisant à sa diminution d'environ 1 885 euros. Ce mécanisme est suspendu par la loi de finances pour et n'affectera donc pas la DGF de la commune en 2023. Si la population de la commune augmente, cette dotation forfaire en fera de même. S'agissant des dotations de péréquation, l'augmentation du potentiel financier de la commune en 2021 et 2022

secrétaire d'État. Je ne suis pas tout à fait convaincu par l'argument de la dotation de compensation par l'agglomération,

Actuellement, les communes et leurs groupements ont le choix entre trois modes de financement du service public d'élimination des déchets : le budget général, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom), la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (Reom). Nous le savons, tous ces modes ne se valent pas pour les collectivités, qui, pour sécuriser le recouvrement, sont de plus en plus nombreuses à opter pour la Teom ou à y revenir. Impôt local assis sur le foncier bâti, la Teom est perçue avec la taxe foncière ; la somme varie en fonction de la valeur locative cadastrale du bien. Elle a pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales. En ce sens, elle diffère de la Reom, dont le montant est calculé en fonction de l'importance du service rendu et de la quantité de déchets produite. Par conséquent, pour les garages, les emplacements de parking et les piscines, locaux par essence non habités et dont l'utilisation ne produit généralement pas d'ordures ménagères, les propriétaires doivent acquitter une contribution si la collectivité chargée de la gestion des déchets fait le choix de la voie fiscale, alors que cette contribution sera nulle dans l'hypothèse d'un financement au service rendu. Par ailleurs, et toujours dans le cadre du choix par la commune de la voie fiscale, des bacs et collectes de déchets sont prévus même pour les locaux par essence non habités, ce qui entraîne un coût non négligeable, Aussi, et dans le souci d'une plus grande équité et d'une rationalisation des coûts, je souhaite savoir si, pour les contribuables dont la propriété n'est pas source de déchets, un ajustement du système Teom pourrait être envisagé.

la Teom pour les collectivités. Monsieur le sénateur, afin d'encourager la réduction et le tri des déchets, une tarification incitative peut être instaurée dans le calcul de la Reom ou de la Teom, par l'introduction d'une part variable qui dépend de la quantité et, éventuellement, de la nature des déchets produits par chaque ménage.

ce plan de fermeture pose un certain nombre de questions aux élus des communes, notamment à ceux de la Loire-Atlantique, département que vous connaissez bien, Je me fais ici même le relais des interrogations du syndicat d'énergie de Loire-Atlantique, le Sydela, sur deux points en particulier. Le premier point concerne tous les services d'urgence et les lignes téléphoniques qui utilisent aujourd'hui le réseau cuivre. Je pense à des infrastructures comme les gymnases, au service de téléalarme pour les personnes âgées, aux ascenseurs

des syndicats. L'arrêt du réseau cuivre est largement souhaitable pour l'ensemble de la filière à de nombreux égards, notamment pour des raisons écologiques, la fibre étant trois fois moins énergivore que le cuivre, ce qui, dans le contexte que nous connaissons, est un enjeu important qu'il faut prendre en compte. Toutefois, madame la sénatrice, comme vous l'avez souligné, la transition du cuivre vers la fibre doit s'accompagner des garanties nécessaires de disponibilité, de qualité et d'abordabilité des services à l'égard de nos concitoyens et des collectivités. Vous avez évoqué des cas très particuliers, comme la téléassistance pour les personnes âgées, qui sont parmi

2015 du programme de fin du réseau téléphonique commuté, le RTC. Les solutions sont donc clairement identifiées aujourd'hui : il s'agit soit de les faire migrer sur la fibre, soit de privilégier l'usage de la technologie GPRS/GSM

lancé en 2013, le plan France Très haut débit, créé pour que l'ensemble des Français aient une connexion internet ultrarapide, fête cette année ses dix ans. Si le déploiement du réseau fibré a incontestablement progressé, les dysfonctionnements sont légion- et c'est peu dire Dans mon département, en Essonne, nous sommes raccordés à 93 %, mais ce chiffre n'est qu'un trompe-l'oeil. Dans la pratique, les interventions sont bâclées, les armoires de connexions dégradées, les déchets de chantiers laissés sur place après travaux, etc. La liste est longue, et non exhaustive. en cause la multiplicité des réseaux et des acteurs ainsi qu'un recours excessif à plusieurs niveaux de sous-traitance. Résultat : en cas de problème, personne n'est responsable de rien et chacun se renvoie la balle Dernièrement encore, mon collègue Grégoire de Lasteyrie, maire de Palaiseau et président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, a été contraint de saisir à deux reprises le gendarme des télécoms, l'Arcep, ou Autorité de régulation Il lui a transmis tous les éléments tendant à caractériser les délits, notamment les dégradations volontaires commises par les sous-traitants opérant sur les infrastructures de réseau. L'Arcep, qui aurait dû dénoncer ces faits au procureur, s'est contentée de répondre que le taux de raccordement du territoire était conforme à la moyenne nationale. Fermez le ban ! C'est donc l'agglomération qui a dû adresser une plainte au procureur de la République d'Évry, conduisant celui-ci à diligenter une enquête judiciaire, laquelle est en cours depuis près de deux ans.

Le deuxième axe porte sur le renforcement des contrôles à la fois par la transmission des opérateurs commerciaux de leurs plannings d'intervention et par la mise en oeuvre de comptes rendus d'intervention permettant le contrôle mutuel entre opérateurs. Le troisième axe porte sur la reprise des infrastructures dégradées, que ce soit au niveau des points de mutualisation ou des réseaux vieillissants ou mal dimensionnés qui nécessitent une reprise globale de l'infrastructure. Plusieurs opérateurs ont déjà notifié un plan de reprise de 1 000 points de mutualisation à l'Arcep, correspondant à 450 000 locaux.

et qu'il s'agit d'une priorité. C'est le cancer le plus fréquent en France et il représente la première cause de décès par cancer chez la femme. Il fait l'objet d'un programme national de dépistage afin d'être détecté précocement et d'en réduire la mortalité, ce dont nous nous félicitons collectivement.

La prise en charge par l'assurance maladie des prothèses capillaires fait apparaître d'importantes lacunes. J'ai été interpellée sur ce sujet par Pascal Beau, directeur d'Espace social européen,

Par ailleurs, la difficulté d'accès aux prothèses composées de cheveux naturels et leur coût contraignent les patientes à un renouvellement régulier des produits prothétiques, contrainte qui accroît le reste à charge. Dans les faits, seulement 40 % des 60 000 personnes éligibles à une prise en charge en bénéficient. La Caisse nationale d'assurance maladie évalue le coût d'une prise en charge totale entre 15 millions et 20 millions d'euros, montant à partager entre le régime obligatoire et les acteurs complémentaires.

La prise en charge des prothèses capillaires a été revue en 2019, afin de prévoir deux catégories : une première sans reste à charge avec un tarif de remboursement de 350 euros ; une seconde avec une prise en charge de 250 euros par l'assurance maladie obligatoire (AMO) et un prix limite de vente à 700 euros.

d'abord de mieux connaître la situation des femmes et de comprendre le phénomène de non-recours. Ensuite, un travail sur les caractéristiques techniques des prothèses sera mené, en lien avec les associations, industriels et distributeurs, pour mieux définir les besoins. Les tarifs et prix limites pourraient alors être revus, afin de mieux calibrer la manière dont l'AMO et, le cas échéant, les complémentaires pourraient prendre en charge ces dispositifs. Cette évaluation permettra ainsi de prévoir de nouvelles modalités de prise en charge des prothèses capillaires

Alertée, l'agence régionale de santé (ARS), en partenariat avec Santé publique France, réalisait alors des études pour comprendre ce phénomène. Ses conclusions, au mois de novembre 2019, confirmaient un nombre de cancers pédiatriques élevé. 2020, après des enquêtes supplémentaires, ces deux agences ont estimé, à la consternation générale, qu'il n'existait pas de foyer de cancers pédiatriques dans ce secteur Plusieurs éléments très concrets nous amènent à douter sérieusement de la qualité et de l'objectivité des recherches menées. En effet, seuls treize cas sur vingt-deux recensés à l'époque ont été retenus, les jeunes de plus de 15 ans en ayant été Des dossiers ont été inversés. Le périmètre géographique retenu était également incompréhensible. Ces constats alimentent un climat de doute et de défiance vis-à-vis des institutions sanitaires.

en arrive à demander à sa maman : « Qui doit vivre ? Qui doit mourir ? », il est urgent d'agir pour faire toute la lumière sur ce phénomène inquiétant, en ordonnant une nouvelle étude beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus cohérente et, surtout, beaucoup plus crédible. La parole ministre déléguée. Monsieur le sénateur, je comprends votre inquiétude et celle des concitoyens de votre département, tout particulièrement les familles touchées par la maladie. Les cancers pédiatriques, qui affectent chaque année environ 2 500 jeunes patients, suscitent légitimement un sentiment d'injustice. la santé et de la prévention est mobilisé et engagé pour mieux prévenir, soigner et accompagner les malades et leurs proches dans ce combat. Si des facteurs liés au mode de vie favorisant le développement des cancers ont été clairement identifiés chez l'adulte, les causes sont rarement identifiées chez l'enfant. La situation du Pays de Retz a été suivie avec grande attention par l'ARS Pays de Loire et Santé publique France, qui ont mené les investigations approfondies et déployé des moyens importants pour déterminer la cause de ces cancers pédiatriques. L'analyse statistique spatiotemporelle n'a pas montré d'anomalie épidémiologique locale, malgré la perception d'un excès de cas par la population. Aussi, une surveillance renforcée des cancers pédiatriques d'une durée de trois ans, soit entre 2020 et 2023, a été engagée dès le mois de

épidémiologique globalement stable, avec une absence de nouveau cas de cancer pédiatrique diagnostiqué depuis le mois de juillet 2021. Les résultats de cette surveillance renforcée ne conduisent donc pas à reconsidérer la décision prise en 2020 de mettre fin aux investigations. La poursuite de cette surveillance renforcée sera évaluée en fin d'année 2023. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des suites de cette décision, monsieur le sénateur. Cette suspicion de cas groupés a mis en exergue les préoccupations de la population en en matière de santé environnementale. Ces dernières trouvent leur traduction concrète dans le contrat local de santé (CLS) de Pornic agglo Pays de Retz, dont le premier axe stratégique vise la promotion d'un environnement favorable à la santé, dans une approche préventive de la lutte contre les cancers.

et de la prévention. Madame la ministre, par cette question, je souhaite appeler votre attention sur les déserts médicaux dentaires. En effet, la difficulté et les inégalités d'accès aux soins bucco-dentaires constituent une réalité sur l'ensemble du territoire français, mais plus encore pour notre ruralité, aujourd'hui bien mise à mal. Bien qu'il existe des mesures incitant notamment les jeunes professionnels de santé à s'installer dans les zones sous-dotées, ces mesures sont insuffisantes, voire inopérantes. L'Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) recommandait déjà en 2021 la formation de 7 265 étudiants en odontologie sur la période 2021-2025. On en est loin ! Vous avez annoncé la création de huit nouvelles facs, mais elles n'ont pas de professeurs. Il y a quelques semaines, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à la consolidation et à la professionnalisation de la formation des internes en médecine générale, afin de lutter contre les déserts médicaux. Ce texte prévoit de faire passer de trois à quatre années la durée du troisième cycle des études de médecine générale. Ainsi, cette quatrième année aurait pu amener les internes à exercer en priorité dans les zones sous-dotées, mais vous avez dévitalisé et rendu cette mesure inopérante dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce dispositif aurait aussi pu être mis en place pour les étudiants en odontologie afin de lutter contre les déserts dentaires. J'imagine que ce n'est pas votre intention, là non plus

Plusieurs départements, notamment le Cantal, sont déjà sinistrés et la démographie, là comme ailleurs, est têtue. Nous ne pouvons attendre que de nouveaux professionnels soient formés en nombre et seulement espérer

ministre déléguée. Monsieur le sénateur, la suppression du traduit la volonté forte du gouvernement d'agir dans une perspective de long terme. Des efforts importants ont été produits afin que les capacités de formation soient portées à la hauteur des objectifs démographiques. Pour la filière d'odontologie, entre 7 000 et 8 000 chirurgiens-dentistes seront formés pour la période 2021-2025, soit une augmentation de 14 % par rapport à la période quinquennale précédente. En outre, le Gouvernement a soutenu, en collaboration avec les collectivités territoriales, la création de huit nouveaux sites universitaires de formation en odontologie. Ces formations ont été installées pour la plupart dès la rentrée universitaire de 2022, à Amiens, Caen, Rouen, Dijon, Besançon, Grenoble, Poitiers et Tours. Ces sites ont été choisis en vue d'orienter les professionnels vers les territoires les plus fragiles du point de vue de la démographie en chirurgiens-dentistes. La création de ces sites de formations s'accompagne d'un renforcement de l'offre de soins dentaires des établissements de santé de ces territoires. De nombreux dispositifs complémentaires ont été mis en place ; je pense au contrat d'engagement de service public (Cesp), dont le nombre de signataires est passé de 76 à 815 entre 2014 et 2021.

Samu (service d'aide médicale urgente) peine à absorber le nombre d'appels au 15 et ne peut répondre comme il le devrait en moins d'une minute. Ne pouvant être orientés dans les délais requis, les patients composent alors le 18, qui, lui-même, est saturé.

de plusieurs facteurs. D'abord, les samedis et dimanches, le Samu est devenu une plateforme de prise de rendez-vous médicaux alors que les médecins ne sont pas présents. Ensuite, on constate une diminution inquiétante du nombre de médecins de permanence. Lorsque la permanence des soins ambulatoires était obligatoire, après vingt heures en semaine et les fins de semaine, le Cher comptait dix médecins de garde ; il n'y en a plus que deux aujourd'hui dans l'ensemble du département. Le constat est alarmant et la situation, déjà inquiétante, risque de devenir gravissime à cause du manque d'opérateurs dans les centres d'appels, du manque de médecins de garde, du manque de médecins généralistes et, aussi, de la saturation de nos services d'urgence. Comment les Comment les Français peuvent-ils avoir accès aux soins au quotidien et, plus dramatique encore, peuvent-ils être sauvés en cas d'urgence vitale si les numéros dédiés ne répondent pas dans les délais ? Madame la ministre, quelles sont les la ministre déléguée. Madame la sénatrice, les tensions que connaissent actuellement les centres d'appels d'urgence proviennent à la fois d'un accroissement structurel de l'activité des Samu, mais également de la situation épidémique hivernale. Plusieurs mesures ont été prises pour aider les centres 15 à y faire face. Les mesures de soutien de la mission flash prévoient un renforcement des équipes de régulation des Samu par le recrutement d'assistants de régulation médicale (ARM) et la revalorisation de la mobilisation des médecins participant à la régulation. Par ailleurs, la mise en place du service d'accès aux soins (SAS) permet de renforcer les centres 15 à travers une régulation médicale commune des appels. La création des SAS ne fait par ailleurs pas obstacle à la mise en place ou au maintien de solutions d'appui par un centre de réception et de traitement des appels d'un autre département. Afin de permettre le déploiement des ARM, un accompagnement financier aux établissements a été mis en oeuvre pour chaque place agréée, la formation des ARM ne relevant pas des formations décentralisées financées par les régions. Il convient de souligner que le ministère a soutenu la démarche de déploiement des centres de formation des ARM, dont le nombre est passé de dix à la fin de 2019 à seize aujourd'hui, soit 641 places places contre 400 auparavant. Le ministère est d'ailleurs actuellement engagé dans une phase de concertation pour faciliter le recrutement d'ARM et adapter leur formation.

Même si la plateforme commune 15-18-112 existe dans le Cher depuis 2005 et démontre toute sa pertinence dans de telles circonstances, les Sdis ne peuvent pas à moyen et à long termes être les supplétifs dans la crise sanitaire. Je rappelle, mais vous le savez, madame la ministre, que nombre de sapeurs-pompiers sont des volontaires et que leurs forces s'épuisent.

(Inserm), ainsi que des universitaires doivent travailler sur les statistiques des décès et des hospitalisations liés au covid-19 selon le statut vaccinal des personnes, toutes causes confondues.

Comment est-ce possible dans un pays comme la France, qui est capable de fournir des données statistiques et médicales très pointues ? À titre de comparaison, le même organisme fournit aux assureurs

Aujourd'hui, madame la ministre, la recherche française n'a accès qu'à des informations partielles, ce qui est totalement insuffisant pour assurer le suivi de l'efficacité de notre politique et de la sécurité sanitaire dans notre pays. Face aux controverses de plus en plus nombreuses, face aux questionnements légitimes, il est urgent que les scientifiques des organismes publics puissent investiguer en toute neutralité, afin de ne pas se limiter aux seules études des laboratoires et des entreprises pharmaceutiques. Pardonnez-moi, madame la ministre, de ne pas comprendre la rétention de ces données, qui sont indispensables pour protéger la santé des Français. La

Le ministère de la santé ne dispose pas des statistiques demandées sous la forme réclamée. Il en est de même concernant d'autres statuts vaccinaux, comme la grippe. Conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où la demande ne portait pas sur des documents existants ni susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, le ministère a demandé à la Cada de déclarer la demande sans objet. Des informations sur le statut vaccinal de toutes les personnes bénéficiaires de soins remboursés par l'assurance maladie, ainsi que leur éventuel décès ou leur hospitalisation, sont disponibles dans le système national des données de santé (SNDS).

ces démarches garantissant la protection des données personnelles, l'intérêt public et la qualité scientifique des projets, conformément à la volonté du Parlement exprimée lors du vote de la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé. Rien ne s'oppose donc à ce que des chercheurs accèdent à ces données pour travailler sur le suivi de l'épidémie, l'efficacité et la sécurité des vaccins et rendent publics leurs résultats, en complément de ce qui existe déjà. Il convient de préciser que les chercheurs de l'Inserm disposent d'un accès permanent et élargi au CNDS les exonérant de ces démarches.

la ministre, j'attire votre attention sur la nécessaire adaptation de la formation des manipulateurs d'électroradiologie médicale (MEM) afin de faciliter leur libre circulation au sein de l'Union européenne. s'agit de trouver une solution pour limiter l'impact des fortes tensions que connaît actuellement cette profession en France. En raison d'une offre de travail insuffisante au regard des besoins de l'offre de soins, les services et les cabinets de radiologie rencontrent des difficultés, parfois aiguës, de recrutements de MEM. Cette situation induit un allongement des délais de rendez-vous pour les patients et complique la réalisation d'examens d'imagerie pour l'ensemble des professionnels. Le nombre d'étudiants français n'a cessé de diminuer en raison à la fois de la baisse du nombre de candidats admis en formation et d'une proportion croissante d'étudiants qui ne terminent pas leurs études. En plus de la pénurie d'étudiants formés, on note également une politique salariale peu attirante dans la spécialité : la profession reste assez méconnue. En Île-de-France, 6 % des postes sont vacants, mais aucune région n'est épargnée. Si l'une des pistes avancées est l'augmentation des effectifs d'étudiants, faciliter la circulation des MEM diplômés de l'Union européenne vers la France vers la France permettrait une amélioration immédiate de la situation dans notre pays. Par ailleurs, les enjeux actuels justifient l'ouverture d'une réflexion sur la création de pratiques avancées

Le passage des instituts de formation sur la plateforme APB en 2017, puis sur Parcoursup, a contribué à une augmentation du nombre d'étudiants. Les concertations menées dans le cadre du Ségur de la santé avec les étudiants des filières paramédicales ont par ailleurs abouti à une revalorisation des indemnités de stage pour certaines formations, dont le diplôme d'État Il convient de rappeler que ce diplôme confère le grade de licence. Pour la circulation à l'échelle de l'Union européenne, la France, comme les autres États membres, reconnaît déjà pour l'accès et l'exercice d'une profession réglementée, comme la profession de MEM, les qualifications acquises dans un autre État membre. Ces qualifications permettent aux titulaires d'exercer cette profession en France. Pour les MEM, comme pour toutes les autres professions ayant des implications en matière de santé publique, l'État membre d'accueil peut toutefois procéder à une vérification des qualifications professionnelles. En cas de différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée par la France de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publique, notre pays peut imposer des mesures de compensation sous la forme d'un stage. Quoi qu'il en soit, qu'il y ait ou non application de mesures de compensation, la reconnaissance des qualifications obtenues dans un autre État membre de l'Union européenne pour la profession de MEM est systématique, conformément au principe de reconnaissance mutuelle.

et de la prévention. Madame la ministre, il a fallu que des agents se perchent sur le toit de l'hôpital Pierre-Janet au Havre et que leurs collègues du centre hospitalier du Rouvray fassent une grève de la faim pour se faire entendre il y a maintenant quatre ans. Faites en sorte, madame la ministre, que nous n'en arrivions pas de nouveau à de telles extrémités ! Les services psychiatriques tentent en effet de tenir le coup face à un véritable raz-de-marée de mal-être, mais cela devient très difficile, tout particulièrement aux urgences. Au Havre, il est ainsi demandé au personnel de gérer la pénurie. L'hôpital manque de médecins, d'infirmiers, de soignants paramédicaux. En outre, seules six chambres individuelles et une chambre de soins intensifs sont disponibles, alors que le nombre d'admissions ne cesse d'augmenter.

2019 au sein des pavillons d'hospitalisation et des urgences psychiatriques. Un pool de nuit a ainsi été constitué. En 2020, 10,7 ETP ont été créés pour renforcer la psychiatrie périnatale. Ils ont aussi permis la mise en service d'une unité thérapeutique pour les auteurs de violences conjugales. 2021 et 2022, une vingtaine de médecins ont également rejoint les rangs du pôle de psychiatrie. En 2021, le contrat territorial de santé mentale a financé, de manière pérenne, à hauteur de plus de 1 million d'euros, la création de 19,8 nouveaux postes médicaux et paramédicaux afin d'améliorer le suivi des patients durant leur parcours de soins.

Ce financement permettra notamment la création de 18 postes supplémentaires, dont 6 en psychiatrie. Les moyens matériels de ce groupement hospitalier seront également considérablement renforcés d'ici à 2030. Ainsi, le GHH prévoit d'investir plus de 36 millions d'euros dans l'infrastructure immobilière de la psychiatrie, d'adapter l'hôtellerie dans les lieux d'accueil et de soins et de mettre

et deux unités d'hospitalisation pour adultes, pour un montant de 25 millions d'euros. Enfin, en 2022, le GHH a perçu 63 millions d'euros de dotation psychiatrie, dont 57,3 millions d'euros de crédits pérennes, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à

et de la prévention. Madame la ministre, j'attire votre attention sur les difficultés croissantes d'accès aux soins hospitaliers dans le Jura. Je vous remercie d'avoir prévu un prochain déplacement dans notre département, tant les hôpitaux de proximité y sont en souffrance. À Saint-Claude, après la fermeture de la maternité et du service de chirurgie hors ambulatoire voilà quatre ans, c'est au tour de l'hôpital de jour pour enfants de fermer ses portes. Service extrahospitalier de pédopsychiatrie construit en 2005 dans un territoire de montagne, il accueillait 195 enfants en 2001, dont 48 s'y rendaient plusieurs fois par semaine pour le suivi de troubles et de pathologies lourdes, comme l'autisme et

et de réanimation (Smur) est fermée, faute de médecins jugés aptes. L'urgentiste à plein temps a été mis à pied pour une question de spécialisation qui ne se posait pas jusqu'à présent.

ministre déléguée. Madame la sénatrice, le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie a en effet été contraint de suspendre temporairement l'accueil de son hôpital de jour de pédopsychiatrie à compter de janvier 2023, le temps de faire face à ses difficultés et de remplacer le praticien référent de cette unité. Je le rappelle, il ne s'agit pas d'une décision de fermeture définitive. Une solution de prise en charge a été proposée par l'établissement à chaque usager, les moyens soignants et les locaux dédiés restant, quant à eux, inchangés. Les autres situations que vous évoquez sont le résultat d'un manque de médecins, ou plus spécifiquement de médecins bénéficiant des diplômes nécessaires pour l'exercice de certaines spécialités, sur votre territoire du Jura.

santé de Bourgogne-Franche-Comté travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires locaux afin de trouver des solutions permettant de répondre localement et à court terme par exemple, à la mise en place, par l'établissement Jura Sud, d'une équipe paramédicale de médecine d'urgence (EPMU), qui sera déployée afin de garantir un temps d'intervention rapide, ainsi qu'une prise en charge par une infirmière diplômée d'État spécifiquement formée à l'urgence et encadrée par des protocoles, en complément et dans l'attente de l'arrivée du Smur. D'autres EPMU seront mises en oeuvre dans les territoires de la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci, madame la ministre. Il est vrai que l'ARS fonctionne bien dans notre territoire, je l'en remercie. Notre population, nos soignants attendent beaucoup de votre visite et nous vous accueillerons avec plaisir. La

Depuis lors, le projet du Gouvernement a changé. Ce dernier souhaite aujourd'hui détruire la tour et construire un nouvel ensemble architectural très imposant. En matière de transition énergétique, madame la ministre, vous ne donnez pas l'exemple ! Cette destruction-reconstruction n'est pas conforme à vos engagements ; une rénovation aurait été plus respectueuse à cet égard. Par ailleurs, il est très regrettable que la maire de Malakoff ait été tenue à l'écart de l'aménagement de cette parcelle. À plusieurs reprises, elle a demandé au Gouvernement de rencontrer les promoteurs du projet pour discuter de son intégration dans la ville

ministre déléguée. Monsieur le sénateur, les ministères chargés des affaires sociales sont engagés dans la démarche de renouvellement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de leur administration centrale, qui vise désormais à regrouper les agents sur trois sites domaniaux en libérant les deux locations privées utilisées actuellement. L'objectif est de rationaliser les occupations, de maîtriser les coûts d'exploitation et de s'inscrire dans une démarche écoresponsable, en réduisant de manière significative la consommation énergétique. Cette démarche de regroupement se traduit par une opération de déconstruction et de reconstruction, qui sera réalisée sur le terrain de l'État anciennement occupé par l'Institut national de la statistique et des études économiques à Malakoff. Attentif aux préoccupations exprimées par les collectivités territoriales, l'État a fait évoluer son projet initial, sans toutefois occulter les besoins fonctionnels et de sécurité des services des ministères qui seront installés sur le site.

La livraison du bâtiment, dont le chantier respectera une charte environnementale et un taux de réemploi des matériaux fixé à 80 %, est envisagée pour le début de l'année 2027, ce qui permettra une installation des services à l'automne 2027.

des bornes de recharge pour les voitures électriques, que l'on peut trouver en particulier dans les stations-service et sur les autoroutes. Lors du salon mondial de l'automobile en France, qui s'est déroulé en octobre dernier, le Président de la République a annoncé un bouclier tarifaire sur toutes les bornes électriques réparties sur notre territoire. Cette idée va dans le sens de la transition énergétique et de l'aide aux familles et aux ménages. Cependant, les prix actuels proposés par les sociétés privées ne sont pas du tout transparents, tant s'en faut. Ils peuvent inclure

et comment le Gouvernement va-t-il prendre les mesures nécessaires à la transparence et à la réglementation des prix de l'électricité sur les bornes de recharge ? À défaut, je crains fort que la conversion à l'énergie électrique dans les transports ne soit un échec. La parole

La recharge ouverte au public des véhicules électriques relève du secteur concurrentiel, dont les tarifs sont librement définis par les opérateurs. Ces tarifs peuvent dépendre des kilowattheures distribués, mais également d'autres facteurs, notamment la rapidité de la recharge. Ainsi, certains opérateurs appliquent des tarifs progressifs au-delà d'un certain temps ou lorsque la recharge est terminée afin d'éviter les « véhicules ventouses » qui bloquent l'accès à la borne et de faciliter l'accès à la recharge d'autres véhicules. Ces tarifs sont transparents et communiqués par les opérateurs de bornes pour chaque station de recharge, mais également par les opérateurs de mobilité dans leur contrat d'abonnement. La tarification réalisée par les opérateurs privés, mais également par les aménageurs publics, inclut naturellement une partie d'amortissement des investissements importants réalisés. Elle prend également en compte les coûts d'exploitation, comme les coûts de supervision ou de maintenance. Elle inclut également les coûts de l'énergie. C'est pourquoi les aménageurs et opérateurs de recharge peuvent, dès lors qu'ils sont éligibles, bénéficier de l'amortisseur électricité mis en place à la fin de l'année 2022. Enfin, des discussions sont en cours à l'échelon européen sur le projet de règlement sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Ce texte a notamment pour ambition de fixer des prix raisonnables,

Je suis satisfait de voir que l'Union européenne va peut-être inciter le gouvernement français à imposer une réelle transparence et une réglementation sur les prix proposés. Nous allons peut-être avancer

Cette mécanique d'incarcération de masse se poursuivra tant que l'on ne se penchera pas sur l'extension du champ pénal et qu'on ne réfléchira pas à une nouvelle ingénierie de la sanction. Les 15 000 nouvelles places promises dans les établissements pénitentiaires ne permettront pas d'améliorer la situation. Elles vont servir à enfermer des gens, mais n'assureront pas le respect du principe de l'encellulement individuel, on le sait.

Il vous en remercie, car elle lui donne l'occasion de réaffirmer le projet porté par le Gouvernement de mettre en oeuvre des conditions de détention plus dignes, mais aussi de meilleures conditions de travail pour nos agents pénitentiaires. Ce sont les objectifs du plan immobilier pénitentiaire, qui prévoit la construction de 15 000 places de prison. La moitié des établissements seront sortis de terre en 2024. Dans votre département, c'est un établissement tout neuf de 600 places qui est en cours de construction à Bordeaux-Gradignan. Il permettra de réduire le taux de surpopulation carcérale de l'établissement actuel. Les travaux ont débuté au mois d'avril 2021 par la construction d'un premier bâtiment, qui sera mis en service au premier trimestre 2024. Un second bâtiment sera mis en service en 2026. Au-delà des nouvelles constructions, le budget alloué aux établissements pénitentiaires s'élève à plus de 130 millions d'euros par an depuis cinq ans, soit le double de ce qui leur était alloué précédemment. Je veux enfin rendre hommage aux surveillants pénitentiaires, troisième force de sécurité intérieure de notre pays, qui font un travail formidable, dans des conditions difficiles. Au-delà des paroles, il y a les actes. C'est pourquoi des mesures sont mises en oeuvre afin de renforcer l'attractivité du métier de surveillant pénitentiaire. La fusion des grades de surveillant et de brigadier entrée en vigueur en 2022 offre aux surveillants un déroulement de carrière plus linéaire, avec une revalorisation indiciaire à la clé. Des revalorisations de l'indemnité pour charges pénitentiaires (ICP) ont également été mises en oeuvre en 2021, en 2022 et en 2023. Enfin, et surtout, le Gouvernement a annoncé une réforme statutaire d'envergure du statut de surveillant dans le cadre de la nouvelle mandature. Elle constituera une réponse efficace au problème d'attractivité des métiers pénitentiaires. La parole

Dans le cadre du Fontenoy du maritime, l'État a prorogé pour trois années supplémentaires ce remboursement, dit, pour les navires battant pavillon français, à l'exclusion, de nouveau, des armateurs exploitant des lignes sous DSP.

l'absence de soutien de l'État dégrade fortement l'attractivité du modèle d'exploitation en DSP. Si le cumul d'aides par exonération et de compensation est contraire aux règles européennes, il semble possible de lever les risques de surcompensation ou de cumul d'aides qui motivent l'exclusion des DSP.

l'entreprise DFDS Seaways, elle a bénéficié du soutien de l'État pour les autres lignes qu'elle opère, à hauteur de 2,8 millions d'euros en 2021 et de 1,5 million d'euros au premier semestre 2022. les entreprises ne bénéficiaient d'aucun soutien. Leur viabilité économique aurait donc pu être très fortement compromise sans cette aide de l'État. Mais le Gouvernement sait à quel point le dumping social fragilise les entreprises. Le secrétaire d'État chargé de la mer travaille sur un panel de